En application de l'article 8 , alinéa 5, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la désignation des vingt-trois membres de la mission d'information sur le thème : « Le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert ». En application de l'article 8 du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (projet n° 100, texte

après l'examen du projet de loi d'urgence relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, je poursuis la feuille de route que je vous ai exposée avec l'examen de ce projet de loi d'urgence relatif est important, car il permettra d'accélérer les procédures administratives de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires dans notre pays, avec deux objectifs : raccourcir de plusieurs années les délais de réalisation de ces projets et contribuer à en réduire le coût pour les consommateurs. Avant d'entrer plus concrètement dans le contenu de ce texte, je souhaite évoquer le contexte dans lequel il s'inscrit. Ce contexte, c'est d'abord celui de l'urgence d'une crise climatique qui menace nos écosystèmes, nos sociétés et l'avenir de nos enfants une crise qui doit nous conduire à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Ce contexte, c'est ensuite celui de la crise énergétique que connaissent l'Europe et une grande partie du monde depuis l'année dernière.

Ces deux crises ont une même origine : notre dépendance aux énergies fossiles pour environ deux tiers de notre consommation finale d'énergie, qu'il s'agisse du gaz, du pétrole et, de manière minoritaire, du charbon. C'est la raison pour laquelle l'ambition du Président de la République et du Gouvernement, conduit par la Première ministre, est que la France devienne le premier grand pays industriel à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles. C'est un impératif pour le climat, bien sûr, mais aussi pour le pouvoir d'achat des Français, pour la capacité d'investissement de nos collectivités et la compétitivité de nos entreprises à long terme, ainsi que, plus profondément, pour notre indépendance politique. Notre stratégie pour sortir des énergies fossiles repose, vous le savez bien, sur quatre grands et indissociables piliers. Il s'agit, d'une part, de la réduction de la consommation d'énergie,

grâce à la mobilisation des entreprises, des collectivités locales et des administrations, ainsi que, plus largement, grâce à la mobilisation des Français, que je veux remercier ici. nous sommes dans les meilleures conditions pour passer cet hiver, mais, surtout, nous continuons à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre alors même que la crise fait rage.

Vous le savez, le Gouvernement fait le choix de la relance de la construction de réacteurs et de la poursuite de l'exploitation des réacteurs en exercice, aussi longtemps que les enjeux de sûreté nous le permettront.

le projet de loi qui nous rassemble aujourd'hui marque une nouvelle phase de notre politique nucléaire, en introduisant un cadre visant à l'accélération du processus des autorisations administratives pour les projets nucléaires. Je veux véritablement y insister : ce texte ce texte ne vise pas à décider de la place de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français, pas plus que des détails du programme de nouveau nucléaire, de la politique en matière de traitement et de recyclage des déchets nucléaires D'autres textes le feront ; d'autres textes l'ont déjà fait. Certaines dispositions isolées, introduites en commission la semaine dernière, concernent ces aspects de la programmation énergétique. Nous aurons l'occasion d'y revenir pendant l'examen des amendements, mais, vous le savez parfaitement, il ne s'agit pas d'un texte de programmation énergétique. En effet, la loi de programmation énergétique doit être précédée d'une grande concertation sur l'avenir de notre mix énergétique, afin de recueillir l'avis des Français sur ce nouveau texte, qui sera soumis au Parlement en 2023. Cette concertation, utile et nécessaire, a commencé en octobre dernier et compte à ce jour plus 25 000 contributions. Elle sera conclue, du 19 au 22 janvier 2023, donc d'ici à la fin de cette semaine, par un forum des jeunesses-

n'en est pas moins très important. En effet, les dispositions prévues préparent l'avenir et sécurisent les délais des décisions que vous pouvez prendre dans les mois qui viennent.

de protection de la biodiversité ou encore de participation du public. Le texte ne modifie ni le processus d'autorisation environnementale ni le processus d'autorisation de création, qui traite des enjeux de sûreté nucléaire. Ces deux autorisations demeurent, tout aussi rigoureuses que par le passé, tout comme les deux enquêtes publiques préalables ou encore le processus de débat public conduit

Il s'applique uniquement aux projets de construction de réacteurs nucléaires localisés à proximité du périmètre de sites nucléaires existants et dont la demande d'autorisation de création est déposée dans les vingt ans suivant la promulgation de la future loi. En effet, vingt ans, c'est le délai qui a été défini par la commission lors de l'examen

ces précisions étant apportées, je tiens maintenant à vous exposer brièvement ce que prévoit ce projet de loi. Afin d'accélérer les projets de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, il rend tout d'abord possible la mise en compatibilité des documents locaux d'urbanisme. En effet, les procédures existantes en matière d'urbanisme sont incompatibles avec la complexité d'un projet de réacteur électronucléaire, et la nécessité de les mettre à jour conduirait à augmenter de plusieurs années la durée de construction. Il permet ensuite de garantir le contrôle de la conformité au respect des règles d'urbanisme, tout en dispensant de permis de construire les installations et les travaux portant sur la création d'un réacteur électronucléaire, ainsi que sur des équipements et installations nécessaires à son exploitation. À compter de l'obtention de la première autorisation environnementale, le texte permet de mener en parallèle l'instruction de l'autorisation de création et les activités relatives aux constructions, aménagements, installations et travaux préalables. En bref, on ne perd pas de temps Ce texte rend également possible la construction de réacteurs nucléaires à proximité des réacteurs existants localisés en bord de mer. C'est une mesure d'importance, puisque, vous le savez, les deux premiers sites envisagés pour l'implantation des deux premières paires de réacteurs sont ceux de Penly et de Gravelines. Au regard de l'intérêt particulier pour la Nation de ces projets nucléaires, ce texte prévoit des mesures de sécurisation de l'accès au foncier, mobilisables en dernier recours et en cas de blocage, en s'inspirant de ce qui existe déjà pour d'autres projets d'ampleurs, comme le projet Iter

Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, cela compte. Proposer un cadre conciliant les impératifs d'accélération et de sécurisation des projets de nouveau nucléaire, ainsi que les plus hautes exigences en matière d'association des parties prenantes, de protection de la biodiversité et de sécurité, voilà l'ambition de ce texte. Ce projet de loi s'insère dans un ensemble de mesures mises en oeuvre visant à poser les rails juridiques, organisationnels, industriels, financiers et procéduraux de la relance d'une politique ambitieuse en matière de nucléaire civil. Il est un maillon d'une stratégie d'ensemble, engagée depuis plusieurs années, pour construire notre indépendance énergétique et mener la bataille du climat en sortant de notre dépendance aux énergies fossiles. Je souhaite conclure en vous indiquant que ce texte est aussi important qu'il est technique. L'enjeu sera d'éviter que de petits grains de sable ne viennent compliquer, ralentir ou fragiliser juridiquement des projets déjà très complexes par nature.

Je tiens à les en remercier. Je salue tout particulièrement le rapporteur Daniel Gremillet et le rapporteur pour avis, Pascal Martin, ainsi que les présidents de commission Sophie Primas et Jean-François Longeot. La parole

mes chers collègues, en 1971, le Président de la République Georges Pompidou s'exprimait en ces termes au sujet du premier plan nucléaire civil : « Il nous appartient de concevoir une politique de l'énergie, politique d'autant plus importante pour la France que nos ressources propres sont modestes. [ ...] Nous avons décidé d'accélérer notre programme d'utilisation de l'énergie nucléaire, considéré comme un facteur important d'indépendance énergétique. ans plus tard, ce constat n'a rien perdu de son acuité. Oui, l'énergie nucléaire est centrale. Et oui, une politique énergétique est indispensable. Or le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, s'il revalorise utilement l'énergie nucléaire, n'offre aucune réponse s'agissant de notre politique énergétique. Je veux le dire solennellement ici : la relance du nucléaire ne peut se résumer à un texte de simplification. Pour réussir, il faut une vision politique cohérente, au-delà de procédures techniques disparates. De plus, le texte manque de perspective et de profondeur, alors qu'il nous est demandé de légiférer jusqu'en 2038, au moins. Le nucléaire de demain ne sera pas celui d'hier. Au-delà de notre indépendance énergétique, il contribuera à notre transition énergétique, car l'enjeu sera d'électrifier pour décarboner, afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Le nucléaire de demain sera confronté à de nouveaux risques, climatiques et numériques. Nos réacteurs devront donc être plus résilients. Le nucléaire de demain sera plus divers. Outre les EPR 2, se développeront des réacteurs de taille ou de technologie différentes, pour réduire les risques et les déchets, ainsi qu'un couplage entre les productions d'électricité et d'hydrogène, utile à l'industrie et aux transports. Enfin, le nucléaire de demain s'inscrira dans une nouvelle société : une société plus décentralisée, où la voix des collectivités et celle des citoyens porteront encore plus, aux côtés de celle de l'État une société plus exigeante aussi, où la sûreté des réacteurs et la gestion des déchets devront être assurées, au-delà de la phase de production. C'est cette vision résolument moderne de l'énergie nucléaire, fondée sur la science et la raison, inscrite dans le monde actuel, ouverte aux technologies futures, que notre commission a souhaité porter, car seule cette vision est à la hauteur des grands défis économiques et énergétiques. Le nucléaire est notre héritage et notre horizon ; sachons le relancer, en tenant compte de ce changement d'époque. Notre commission est très attachée à l'énergie nucléaire. Nous l'avons démontré dans nos travaux législatifs, avant et bien souvent contre le Gouvernement. Ce ne fut pas simple de décaler de dix ans le calendrier de fermeture des réacteurs dans le cadre de la loi Énergie-climat de 2019. Ce ne fut pas simple, non plus, de conditionner toute autre fermeture à la prise en compte de ses conséquences sur notre sûreté, notre approvisionnement et nos émissions lors de la loi Climat et résilience de 2021.

Lors de mes travaux préalables, j'ai entendu une centaine de personnalités au cours d'une cinquantaine d'auditions. Je remercie vivement le rapporteur pour avis, Pascal Martin, des excellentes relations de travail que nous avons nouées ; elles nous ont permis d'organiser des auditions communes et de présenter des rédactions communes. Cela confère au Sénat une voix forte et unique sur ce sujet essentiel. Je retiens de ces travaux préalables l'existence d'un large consensus autour de l'objectif du texte, mais aussi de lourdes critiques portant sur la méthode. S'agissant de son objectif, le texte doit permettre d'accélérer la construction de nouveaux réacteurs : d'une part, certaines procédures sont simplifiées, notamment en matière d'urbanisme, de construction ou d'expropriation ; d'autre part, certains actes voient leur nombre réduit et sont élevés au rang du décret,

le Gouvernement omet les consultations en cours, la Commission nationale du débat public ayant été chargée du débat portant sur l'évolution du mix énergétique et sur le programme du nouveau nucléaire, dont le site de Penly. Enfin, le Gouvernement se focalise sur la simplification, éludant les questions cruciales de la révision de la planification énergétique, de la décision de construction des réacteurs, ainsi que des moyens financiers et humains nécessaires, avec en filigrane le devenir de la régulation du nucléaire et du groupe EDF. Surtout, ce texte ne doit pas faire oublier la responsabilité du Gouvernement dans le déclin de la filière du nucléaire. Jusqu'en 2022 et le tournant du discours de Belfort, il a appliqué une politique d'attrition du nucléaire existant et d'indécision s'agissant du nouveau nucléaire. Or, pour notre commission, il faut renverser la tendance ; il faut non pas se limiter aux annonces du discours de Belfort, mais construire davantage d'EPR 2. Dans ce contexte, j'ai fait adopter une quarantaine d'amendements en commission, afin de une quarantaine d'amendements en commission, afin de compléter le texte selon quatre axes majeurs. Le premier axe vise à en combler les angles morts. À cette fin, j'ai proposé d'allonger à vingt ans la durée des mesures de simplification et d'y intégrer, aux côtés des EPR 2, les projets de SMR et d'hydrogène. J'ai également voulu clarifier la notion de « proximité immédiate », selon les préconisations de l'Association des maires de France J'ai aussi prévu que l'État rende compte au Parlement de la mise en oeuvre des mesures et des chantiers, afin que celui-ci soit informé sans omission des éventuels dépassements de délais et de coûts. L'État devra nous indiquer les sites retenus par EDF. Une clause de rendez-vous permettra d'inclure de nouveaux sites et de nouvelles technologies. De plus, j'ai proposé de réviser la planification énergétique, en levant les verrous issus de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Il faut abroger l'objectif de réduction à 50 % de l'énergie nucléaire d'ici à 2035 et le plafonnement à 63,2 gigawatts des autorisations d'exploitation.

et le climat, attendue d'ici à juillet prochain, acte la construction des nouveaux EPR 2 et SMR d'ici à 2050 et précise les moyens financiers et humains requis. Le deuxième axe vise à garantir la sûreté et la sécurité. Dans cette perspective, j'ai proposé d'intégrer la résilience au changement climatique dans la démonstration de sûreté des réacteurs, tant de leur autorisation que de leur réexamen, ainsi que la cyberrésilience à la protection des réacteurs contre les actes de malveillance. J'ai aussi voulu conditionner l'octroi des concessions d'utilisation du domaine public maritime à la prise en compte des risques de submersion, d'inondation et de recul du trait de côte. ailleurs, j'ai entendu maintenir le rapport quinquennal sur la sûreté, encadrer le recours à la simple déclaration préalable dans le cadre du réexamen des réacteurs et clarifier les délais de la procédure de mise à l'arrêt définitif. Enfin, j'ai voulu moderniser le fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire, en renforçant les attributions de sa commission des sanctions et en actualisant les règles, les évaluations, les prescriptions ou les infractions applicables. Le troisième axe vise à associer les collectivités territoriales et le public. Pour ce faire, j'ai souhaité garantir que les réacteurs ne puissent être qualifiés d'intérêt général qu'après la tenue du débat public. J'ai aussi voulu que les collectivités puissent amorcer un dialogue avec l'État s'agissant de la modification de leurs documents d'urbanisme.

et dernier axe vise à renforcer la sécurité juridique des procédures. Tout d'abord, j'ai proposé que les travaux pouvant être anticipés le soient, aux frais et aux risques de l'exploitant et après information du public. J'ai également voulu qu'un décret détermine ces travaux après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). J'ai aussi garanti le contenu de l'étude d'impact, les modalités de l'enquête

ailleurs, j'ai proposé de réduire à six ans le délai de la procédure d'expropriation, d'en exclure les ouvrages de raccordement et les équipements de fonctionnement, ainsi que de prévoir des garanties, notamment de relogement des habitants ou d'indemnisation des professionnels. Enfin, j'ai ajouté deux procédures manquantes

entre effort de simplification et exigences renforcées de sûreté et de sécurité. Je forme le voeu que ce texte contribue à la relance du nucléaire. Dans la crise énergétique que nous traversons, l'énergie nucléaire est un atout pour offrir un coût de l'électricité attractif. Il faut

la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, au nom de laquelle je m'exprime aujourd'hui, salue le signal sans équivoque que constitue le texte soumis à l'examen du Sénat. Après de trop nombreuses années d'atermoiements, ayant conduit à un délaissement de la filière nucléaire, préjudiciable pour le climat, mais aussi pour la préservation de notre souveraineté, la nouvelle impulsion énergétique et industrielle est bienvenue. Elle est même indispensable au maintien de la France à sa place de numéro un de l'électricité décarbonée et au soutien de l'électrification des usages prévue par la stratégie nationale bas-carbone, à une production pilotable, en parallèle du développement des énergies renouvelables et de la réduction massive de notre consommation énergétique. Notre commission a toutefois regretté la méthode consistant à aborder le particulier avant le cadre général il eût été préférable, pour la clarté des débats politiques, de définir au préalable les objectifs de la politique énergétique dans le cadre de la loi de programmation sur l'énergie et le climat, qui doit être adoptée au Parlement dans le courant de l'année 2023. En dépit des réserves et des remarques que je vous présenterai ici succinctement, notre commission a donné un avis favorable au présent projet de loi. Compte tenu du champ très restreint du texte, de sa grande technicité et du calendrier des consultations actuellement à l'oeuvre concernant les projets des six premiers EPR 2, ainsi que de l'élaboration de la stratégie française pour l'énergie et le climat, notre commission a souhaité apporter au texte des ajustements essentiellement juridiques, avec un double objectif : premièrement, améliorer la sécurité juridique et la lisibilité du texte, afin de limiter les risques contentieux qui affaibliraient la relance souhaitée du nucléaire français ; deuxièmement, encadrer les marges laissées au pouvoir réglementaire. du premier objectif, notre préoccupation principale a été de mieux définir la notion de proximité immédiate, telle qu'elle est proposée par le Gouvernement à l'article 1. Nous pensons que cette notion pourrait correspondre à toute implantation ne nécessitant pas de modification de la zone d'application et du périmètre du plan particulier d'intervention, aussi appelé PPI, des centrales nucléaires existantes. À l'article 4, nous avons également souhaité définir plus précisément par voie réglementaire les bâtiments sensibles dont la construction ne pourra être entreprise qu'après la délivrance de l'autorisation de création et ceux, à moindres enjeux de sûreté, qui pourront commencer dès l'octroi de l'autorisation environnementale. objectif visant à encadrer les marges laissées au pouvoir réglementaire, notre commission a souhaité que ce dernier soit contraint d'ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, dès lors que l'absence de volonté ainsi que l'incapacité de l'exploitant de remettre son installation en service dans des délais raisonnables sont constatées par la puissance publique. Cette option nous semblait équilibrée et offrait une opportune valeur ajoutée : elle évitait les instructions inutiles, comme le souhaitent les auteurs du projet de loi, sans pour autant affaiblir le principe d'un démantèlement des installations, le plus tôt possible, après leur arrêt. Elle n'a pas été retenue lors de nos débats en commission. Avant de conclure, j'aimerais rappeler que ce projet de loi, aussi bienvenu soit-il, aura un impact limité sur la relance du nucléaire français l'accélération des procédures et la réduction du risque contentieux ne constituent que des leviers mineurs pour s'assurer du développement dans les délais souhaités d'un nouveau parc et de la prolongation du parc existant dans les conditions de sûreté adaptées.

et, d'autre part, à assurer une acceptabilité locale et nationale autour de la relance du nucléaire. En résumé, il conviendra en 2023 de donner une visibilité suffisante aux acteurs du nucléaire l'anticipation, indispensable à la fois à la montée en compétences de la filière et à l'acceptabilité du nouveau programme, constitue sans aucun doute la meilleure réponse aux défis qui s'annoncent pour le nucléaire français. Nous passons à la discussion nucléaire français. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

selon une approche rationnelle, est évidente : c'est non, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en mettant ce projet de loi à l'ordre du jour du Parlement, le Gouvernement ne respecte pas le débat démocratique qui a lieu en ce moment même- nous sommes là dans le droit fil de l'histoire du nucléaire.

Ce projet arrive également avant les débats qui doivent se tenir autour de la future loi quinquennale de programmation sur l'énergie et le climat, dont doivent découler la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas-carbone. C'est à l'issue de ces débats, et évidemment pas avant, que sera défini notre mix énergétique, et je note que, sur ce point, nous sommes en accord avec le rapporteur.

Demander aux parlementaires de voter un projet de loi actant une relance du nucléaire avant cette loi de programmation, alors qu'aucune obligation légale ou réglementaire ne l'impose, nous paraît largement prématuré et profondément anti-démocratique. Quel est l'objectif, sinon mettre les acteurs concernés, ainsi que nos concitoyens, devant le fait accompli ? Toutes les garanties doivent être apportées pour que ces choix politiques soient pris dans le respect du Parlement et de nos concitoyens, et non décidés unilatéralement par le chef de l'État, à Belfort. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'oppose au fondement même du projet : la relance du nucléaire. Nous ne pouvons que nous y opposer, même si nous sommes lucides sur le fait de devoir encore, hélas ! composer avec le nucléaire existant un certain temps. Depuis des années, en effet, l'inaction est de mise sur l'efficacité et la sobriété, et le rythme de développement des énergies renouvelables n'a pas été respecté. Il n'est pas acceptable de relancer des activités nucléaires polluantes et dangereuses qui nous engagent pour au moins un siècle, alors que les menaces de tous ordres, en particulier les bouleversements climatiques, vont accroître de façon considérable les risques encourus par cette filière. Qui peut vraiment prédire le climat et l'état de la planète en 2050, alors qu'il y a déjà d'énormes incertitudes sur les cinq ans à venir ? Ce n'est pas acceptable, d'autant que des solutions alternatives totalement crédibles, non dangereuses, plus rapides à mettre en oeuvre et bien moins chères sont à portée de main. Nous tenons en premier lieu à souligner l'incohérence de l'objectif affiché dans l'exposé des motifs quant à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

du climat, classe le nucléaire loin derrière les énergies renouvelables et les économies d'énergie, au regard des objectifs de développement durable qu'il a établis, en prenant en compte les coûts élevés, la nécessité d'un soutien public très important, l'enjeu de la gestion des déchets, les impacts sur les ressources en eau, la pollution liée aux mines d'uranium, le risque de prolifération, etc. Nous ne pouvons exposer la question du nucléaire sans parler des enjeux de sûreté. Les impacts des accidents nucléaires survenus dans le passé perdurent. Ainsi, trente-six ans après l'accident de Tchernobyl, des territoires entiers restent contaminés. Il ne suffit pas de minimiser les faits d'une manière mensongère dans une bande dessinée pour que cela devienne réalité ! Il faudra des siècles pour que la radioactivité disparaisse des sols. À Fukushima, il faut continuer à refroidir le combustible. Plus d'un million de tonnes d'eau contaminée restent présentes sur le site.

Selon Gregory Jaczko, ancien président de l'Autorité de sûreté nucléaire américaine, les accidents nucléaires graves sont inéluctables. Le nucléaire est un malade chronique, qu'il faut surveiller sans cesse en temps de paix. Mais il faut ajouter à cette maladie une vulnérabilité intrinsèque face aux agressions extérieures, ce qui en fait une énergie profondément dangereuse. Nous pouvons le constater encore aujourd'hui avec la situation gravissime autour de la centrale de Zaporijia, en Ukraine.

Certains associent facilement nucléaire et souveraineté, mais depuis quand « nucléaire » rime-t-il avec « indépendance énergétique » ? Nos 210 mines ont produit en totalité l'équivalent de dix ans de consommation. Elles sont toutes fermées depuis vingt ans. Aujourd'hui, 100 % du combustible est importé. Ces importations se font au prix de compromissions avec certains régimes autoritaires et au mépris de la santé des populations locales. Au Niger, par exemple, l'extraction d'uranium suscite des poussières radioactives, empoisonne l'eau et la nourriture et affecte la santé des habitants. Quant au coût du démantèlement des centrales en fin de vie, sur ce sujet comme sur d'autres, EDF avance des chiffres totalement fantaisistes, déconnectés des réalités.

Pour les moins radioactifs, issus des démantèlements, la solution avancée semble être la dissémination, la dilution dans l'environnement. Tout cela a et aura des coûts faramineux, et c'est bien le contribuable qui devra mettre la main au portefeuille- une habitude pour le nucléaire où va-t-on vraiment gagner du temps avec ce projet de loi ? Ce ne sont pas les procédures administratives en matière d'urbanisme ou de droit de l'environnement qui freinent le déploiement du nucléaire, comme le laisse croire ce texte. Cette analyse simpliste ne permet pas de poser les vraies questions sur les défaillances et les contraintes structurelles de l'énergie atomique. Il faut plutôt chercher dans les domaines du travail de conception, des études détaillées, de l'instruction technique. À tout cela s'ajoute l'absence de compétences, qui suscite des malfaçons en cascade. J'en viens au fleuron, l'EPR, la définition même de ce que l'on appelle un fiasco industriel et économique, cause au mois de juillet 2020 par la Cour des comptes elle-même, au travers d'un rapport extrêmement sévère sur la filière. Ce rapport revient sur la longue liste des problèmes responsables des retards interminables et du surcoût du chantier de Flamanville, ainsi que des autres réacteurs en construction de par le monde. Surtout, la Cour des comptes met en doute l'opportunité de relancer un nouveau parc nucléaire, appelant l'État à se demander si d'autres options de production d'électricité ne sont pas plus pertinentes et moins chères. en effet, est aussi un gouffre financier. Ce qui pourrait seulement interroger devient proprement scandaleux lorsque le coût estimé pour Flamanville atteint désormais près de 20 milliards

le retour d'expérience sur ce fiasco de l'EPR est incomplet. Refuser de tirer les leçons de ce chantier catastrophique avant d'engager la France dans des projets de nouveaux réacteurs, qui connaîtront très probablement à leur tour retards, surcoûts et malfaçons, n'est pas acceptable. Décider le lancement de ces projets revient à mépriser la démocratie, la sûreté et les générations futures, qui devront porter le poids de ces nouveaux boulets à leurs pieds. Alors que cet échec industriel et économique n'est plus à démontrer, est-il opportun de remettre une pièce dans la machine ? Le Gouvernement, comme l'administration, s'arc-boute sur des schémas du XX siècle- on a précédemment évoqué le président Pompidou. Il reste habité par cette mystique qui veut que la grandeur de la France passe nécessairement par une industrie nucléaire triomphante, à l'énergie prétendument peu chère et abondante. Se lancer sur cette trajectoire de construction de nouveaux réacteurs, c'est mettre quasiment tous nos oeufs dans le même panier, avec toutes les incertitudes sur les délais, les coûts et les garanties de sécurité que cela comporte. De tels investissements asphyxient tous les autres besoins de financement pour la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. C'est proprement irresponsable Pour conclure, les propositions des sénateurs et sénatrices écologistes sont claires. Les économies d'énergie couplées à une rapide montée en puissance des énergies renouvelables, une production tout à la fois décentralisée et en réseau : voilà la vraie transition énergétique que nous défendons

Quel est l'avis de la commission ?

s'est assurée que les consultations avaient bien été effectuées, notamment celles du Conseil national de la transition écologique, du Conseil national d'évaluation des normes et de la mission interministérielle de l'eau.

se poursuivent sous l'égide de la Commission nationale du débat public. J'ajoute que notre commission est très sensible à la question de la participation du public. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu lors de nos travaux, d'une part, que la qualification de projet

que nous ayons des réacteurs nucléaires en 2035 ou 2037, ce qui est l'objectif du Gouvernement. En d'autres termes, nous ne confondons pas vitesse et précipitation. Nous sommes

Nous n'examinons pas aujourd'hui le texte du Gouvernement, dont l'objectif était d'anticiper sur les plans administratif et juridique les décisions à venir,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes ici une majorité à être d'accord pour simplifier et alléger le carcan normatif pesant sur la construction de nouvelles centrales nucléaires et l'entretien du parc existant. Cependant, nous ne saurions réduire le débat sur ce projet de loi à de simples allègements administratifs, sans évoquer la vision et le cap de notre politique énergétique, si tant est qu'il en existe encore un. La temporalité de l'examen de ce texte est tout d'abord doublement anachronique. Nous sommes encore soumis à la mauvaise trajectoire de la précédente

la fermeture de quatorze réacteurs nucléaires d'ici à 2035, pour passer la part du nucléaire de 80 % à 50 % dans notre mix énergétique national. Les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim ont ainsi été fermés en 2020 après quarante-trois ans de fonctionnement, soit la moitié de la durée de vie de certaines centrales aux États-Unis, et alors que nous avons une ingénierie de pointe en la matière. Vous êtes, madame la ministre, pour le départ à la retraite à 64 ans pour tous, sauf pour les réacteurs nucléaires ! Puisque le présent texte prévoit désormais le départ à la retraite des réacteurs au-delà de 60 ans, il serait incompréhensible de ne pas revenir sur cette décision. Cette centrale, en effet, ne présentait aucun dysfonctionnement mettant en cause la sûreté de l'installation. À cette problématique s'ajoute celle, d'ordre juridique, qui consiste à savoir si l'on peut définir une stratégie souveraine, indépendamment de celle que fixent les institutions européennes, sous le regard attentif et la main interventionniste de l'Allemagne. Aujourd'hui, notre filière nucléaire est la première victime des choix de Bruxelles, que vous appliquez avec le zèle qui vous caractérise. Dès lors, oui, je ferai tout pour actionner les faibles leviers qui sont les nôtres en faveur de la prolongation des centrales existantes et la construction d'EPR de nouvelle génération et de petits réacteurs modulaires. Mais, non, je ne participerai pas à l'enthousiasme communicationnel autour de ce tout petit texte rédigé à la hâte, car je suis chaque jour aux côtés des Français qui voient leur facture énergétique exploser en raison de vos choix désastreux. Je suis aux côtés des artisans et des entreprises précarisés, non pas à cause de la guerre en Ukraine, mais à cause de vos renoncements sur la filière nucléaire, notamment l'abandon du projet Astrid (), après celui de Superphénix. de Superphénix. Je suis aux côtés des maires qui voient leur budget rabougri, obérant le développement de leur commune. Les événements du dernier week-end en Allemagne sont l'image parfaite de ce que nous ne voulons pas voir chez nous une guerre sociale, des villages détruits pour des mines et d'ignobles éoliennes qui s'étendent avec un appétit sans fin. C'est pourtant ce qui se profile avec la réouverture du site de Saint-Avold

les inquiétudes exprimées à la fin de l'année 2022 et les plans de délestage annoncés dans la presse constituent une piqûre de rappel- s'il en fallait une ! -quant à la vulnérabilité de notre approvisionnement en énergie. Nous échapperons probablement aux coupures cet hiver, grâce aux efforts des Français, qui réduisent leur consommation d'énergie, au redémarrage de nombreux réacteurs durant le mois en cours et aux températures clémentes des trois dernières semaines. Mais pour combien de temps ?

Nous sommes donc au tournant de la sortie progressive de l'ère des énergies fossiles, sortie qui, au regard du retard pris, s'annonce abrupte. Elle implique notamment de décarboner tous les secteurs, à commencer par celui de l'énergie, et ainsi de doubler notre production d'électricité.

Tous les scénarios présentent de fortes incertitudes quant à la disponibilité des technologies, au contexte social, géopolitique et macroéconomique, aux besoins en formation ou au financement. Dans tous les cas, le groupe RDSE soutient de longue date un mix énergétique diversifié, combinant nucléaire, énergies renouvelables (EnR) et hydrogène, afin de garantir la stabilité du système électrique, lequel doit demeurer pilotable.

Aussi, il faut aller vite et relancer un nouveau programme nucléaire. Après l'examen d'un projet de loi consacré à l'accélération des énergies renouvelables, on ne peut que se réjouir du retour en grâce de l'atome, à la fois en France et sur la scène internationale. En pariant sur le nucléaire, en confirmant ses choix historiques, qui lui ont permis de produire une électricité largement décarbonée, la France ne fait pas cavalier seul. Cependant, le temps long de la construction des réacteurs implique de prendre dès à présent pour compter sur une première mise en service en 2035 et un parc de quatorze EPR en 2050. Cette accélération ne doit pourtant pas être synonyme d'escamotage de la démocratie participative ou représentative ou encore des règles de sécurité et de sûreté. C'est bien cela que garantit ce projet de loi, en facilitant la construction de nouveaux réacteurs sur les sites existants ou dans leur proximité immédiate, afin de s'assurer de l'acceptabilité des projets.

J'ai déposé un amendement visant à ce que les études de faisabilité concernant la construction de ces réacteurs soient rendues dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, afin de donner de la visibilité à ce territoire qui dispose de tous les atouts pour les recevoir. recevoir. Examiné en commission, celui-ci a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. J'en prends acte. Nous le savons, les défis de la filière nucléaire ne reposent pas seulement sur les démarches administratives. Le projet de loi ne produira qu'un gain de temps mineur, certes non négligeable : un raccourcissement des délais de cinquante-six mois, selon le rapporteur au fond. Des obstacles plus importants nous attendent, qui sont de plusieurs ordres : délais industriels ; solutions à trouver aux problèmes de construction apparus sur le chantier de Flamanville ; formation et maintien des compétences ; sécurité d'approvisionnement en uranium dans un contexte géopolitique

Fin 2022, au moment même où, plus que jamais, nous avions besoin de cette source d'énergie pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, la moitié de nos réacteurs était encore à l'arrêt, symptôme apparent d'une situation moins visible, mais structurellement grave. En réalité, jusqu'au discours de Belfort, tenu fort opportunément à la toute fin du précédent quinquennat, à revers de la politique menée jusque-là, le Gouvernement a totalement délaissé la filière du nucléaire. Il est même allé, ne l'oublions pas, jusqu'à céder les capacités de production de turbines nucléaires d'Alstom, dans une bataille géoéconomique et géopolitique épique.

pour soutenir notre économie, sans aucun investissement à la clé ? 50 milliards d'euros d'eau sur le sable en un an, contre 1,5 milliard d'euros pour semer l'énergie de demain ... Le compte n'y est pas

sauf motif de sûreté, en l'absence d'étude d'impact sur la sécurité de notre approvisionnement énergétique et sur les émissions de gaz à effet de serre. Je me souviens

Surtout, ce manque d'ambition vis-à-vis du nucléaire a asphyxié une filière qui, se croyant en déclin, n'a plus attiré ni les talents en nombre suffisant ni le volume d'investissements nécessaire. Tout à fait

d'oublier les conséquences délétères de cette politique de l'abandon. RTE n'a-t-il pas placé la France en situation de « vigilance particulière » jusqu'en 2024 en matière de sécurité d'approvisionnement ? L'Ademe évoque, quant à elle, une « érosion tendancielle » de la production nucléaire depuis dix ans, un système électrique « sans marge ». Il est donc urgent d'agir, au-delà du texte de simplification proposé. Le Gouvernement doit lancer la construction effective des réacteurs, les six annoncés

Enfin, et surtout, la recherche et le développement doivent être soutenus pour renforcer nos capacités d'innovation et d'attractivité, notamment en ce qui concerne les réacteurs de quatrième génération

non disponibles sur notre territoire se trouve dans la recherche, dans le bouillonnement de l'innovation, dans l'optimisation et dans le recyclage de ces matériaux. Le nucléaire est une énergie qui offre aux Français et à nos entreprises un coût d'électricité inférieur à celui que

par ailleurs, l'une des conditions du développement de l'hydrogène, qui pourrait être produit à grande échelle à partir de l'électricité de nos réacteurs. Oui, madame la ministre, notre commission a transformé ce texte technique en affirmation d'une volonté politique pour réussir enfin la relance de l'énergie nucléaire, pour donner ce signal tant attendu depuis plus de dix ans. Au-delà de la simplification normative, nous avons souhaité dessiner une véritable trajectoire de relance, pour un nucléaire plus abondant, plus sûr, plus rapide et plus innovant. Nous ne pouvions nous résoudre à indiquer, comme vous le faisiez dans le texte d'origine, qu'il faut « accélérer l'installation de nouveaux réacteurs, accélérer la prolongation des centrales actuelles », tout en actant les prochaines fermetures de douze anciens réacteurs actifs. d'une contradiction flagrante ! Cette coordination juridique d'une cohérence politique et de l'affirmation d'une ambition énergétique devait être opérée

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un grand Lorrain, Pierre Messmer, alors Premier ministre, déclarait en 1974 : « Notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Malheureusement, trop d'années d'inaction, d'hésitation, d'atermoiements et de renoncements, trop de choix stratégiques souvent guidés par des opportunités politiques court-termistes, puis sacrifiés au profit de coalitions de circonstances, ont fragilisé ce fleuron industriel.

Ce texte est nécessaire, car il est urgent d'agir pour remettre en marche notre filière nucléaire. Il comporte deux grands volets. Le premier volet porte sur la simplification des procédures réglementaires et administratives liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites existants le second a trait au fonctionnement des installations. Ce projet de loi pose en définitive le cadre d'une accélération procédurale. Je veux saluer le travail de précision effectué par la commission des affaires économiques sur ce texte

une orfèvre en matière de déplanification énergétique ! Quelle absence de réalisme, quel manque de vision ! Ce texte renforce utilement la place des collectivités territoriales.

Le nucléaire porte le triple objectif de souveraineté énergétique, d'indépendance de la Nation et de décarbonation de nos modes de vie. Nous devons néanmoins apprendre de nos échecs passés,

accueille le projet Cigéo de stockage des déchets nucléaires français. Madame la ministre, je sais que vous êtes particulièrement engagée sur ce dossier. Ce projet, assis sur le travail d'un laboratoire expérimental, d'un laboratoire expérimental, vise à sécuriser durablement les déchets. Il concourt pleinement à la crédibilité et à l'acceptation du nucléaire, au travers d'une maîtrise totale de la filière. Il s'inscrit dans un temps très long et laisse la porte ouverte aux innovations futures. Cela doit nous inspirer. Madame la ministre, le chemin est encore long et les défis très nombreux. Cependant, les derniers résultats concernant la fusion sont très encourageants. Ce texte constitue une première étape pour la relance du nucléaire, laquelle est absolument nécessaire, car elle conditionne notre avenir industriel, économique et social. Fort de ces constats, et prêt à prendre toute sa part dans ce nouveau défi, le groupe Les Indépendants - République et

J'ai un peu hésité sur la qualification de cette aventure industrielle unique au monde : « épopée », « odyssée » ? ... Finalement, « conte de fées » me semble convenir le mieux, tant cette histoire fait appel au merveilleux merveille technologique, une merveille économique et, chapitre plus récent, sous les augures du mage Jancovici, une merveille écologique. Tout est dit, mais il reste de petits « mais Les vrais amateurs le savent bien, de Charles Perrault aux frères Grimm, la fin d'un conte est souvent tragique et ne ressemble pas toujours à un dessin animé de Walt Disney. La faillite retentissante d'Areva en est une malheureuse illustration dans le conte de fées nucléaire français.

Peu importe, tout cela est du passé, car, de la brume normande, surgit l'EPR flambant neuf de Flamanville, dont les électrons se déversent déjà en masse sur l'Ouest breton Ah, on m'informe qu'une vilaine sorcière mal intentionnée- peut-être Dominique Voynet ? -l'a transformé en Belle au bois dormant. Je sais toutefois que, dans cet hémicycle, se trouvent de valeureux guerriers, prêts à traverser les landes du Cotentin pour réveiller la belle endormie En outre, pas d'inquiétude, je suis en mesure de vous informer que nos ingénieurs français avaient découvert avant tout le monde la formule du béton du forum romain, l'un des secrets les mieux gardés de l'Antiquité,

Empêtrée dans un dogme libéral suranné, nourrie de calculs à courte vue sur les prix de revient du mégawattheure, la totalité de nos voisins n'est pas capable de financer pendant autant d'années une machine qui ne fonctionne jamais.

Nous allons battre- nous pouvons en être fiers, c'est le génie français ! -le record du monde du prix le plus élevé du mégawattheure issu d'une machinerie industrielle de production électrique.

Sommes-nous encore dans un conte de fées ou dans une fable ? J'hésite. Sans perdre le fil littéraire de mon propos, et au risque de verser dans une sécheresse technocratique qui ne me sied guère,

Reste la merveille écologique, que nul ne peut contester : une production décarbonée et infinie. Enfin, ce qui est infini, c'est surtout la durée de vie des déchets, pour lesquels nous ne disposons toujours pas de solution, sinon creuser des trous.

soeur Anne- de Bretagne -ne voit toujours rien venir à Brennilis, où l'enveloppe du coeur n'a toujours pas été percée, à l'inverse du reliquaire. Heureusement, Catherine Deneuve n'a pas encore eu la peau de l'âne qui paye le budget de l'État, car le démantèlement de nos vieilles centrales n'est, je le rappelle, toujours pas financé

Deux facteurs principalement expliquent cette faible disponibilité du nucléaire : les opérations de maintenance classique et, surtout, un problème de fissuration, dit de corrosion sous contrainte, un mal mystérieux qui menace des tuyauteries de secours destinées au refroidissement

Le problème générique sur les réacteurs a été pris très au sérieux et, sur les dix chantiers ouverts, six sont désormais terminés. Ainsi, en ce milieu d'hiver, seuls douze réacteurs sont à l'arrêt, contre plus de trente au sortir de l'été. Le pire est donc passé, lorsque l'on sait que le pays a dû se résoudre, en 2022, à importer plus d'électricité qu'il n'en a exportée- une première en quarante ans. Cette année difficile pour le parc nucléaire doit nous conduire à nous interroger sur ce que nous souhaitons pour assurer notre indépendance énergétique. Face au dérèglement climatique- l'année 2022 est la plus chaude jamais mesurée en France, afin d'assurer une sécurité d'approvisionnement, ce gouvernement a choisi de construire sa stratégie énergétique autour de deux axes : les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. nucléaire. Notre groupe se réjouit que le Gouvernement ait choisi de reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France, avec la construction de six EPR 2 et le lancement d'études sur la construction de huit EPR 2 additionnels. une fois ce cadre politique posé, vient le temps essentiel de la concertation, un moment démocratique indispensable pour recueillir l'avis des citoyens sur les orientations de la politique énergétique française et permettre à chacun de s'exprimer sur les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de transition énergétique. Cette concertation nationale a commencé le 20 octobre et prendra fin demain, le 18 janvier.

En attendant, plutôt que d'être dans la passivité, notre gouvernement a choisi d'agir et d'accélérer, et nous nous en félicitons. Tel est l'objet de ce projet de loi,

je souhaite ardemment que le site du Tricastin puisse accueillir deux nouveaux réacteurs ; quelque 135 hectares y sont d'ores et déjà disponibles pour donner une nouvelle impulsion économique et industrielle à notre région.

propose ainsi de dispenser de permis de construire les installations et les travaux de création d'un réacteur nucléaire. La construction de réacteurs électronucléaires induit en effet des contraintes que le permis de construire ne permet pas d'appréhender dans leur intégralité. intégralité. Il permet aussi de démarrer certains travaux dès l'obtention d'une autorisation environnementale. Cela concerne des activités qui ne revêtent aucun caractère sensible, comme les travaux de terrassement ou de construction des bureaux, voire la construction de clôtures et de parkings nécessaires au chantier. de la centrale de Penly, il est proposé de construire de nouveaux réacteurs nucléaires en bord de mer. La particularité de cette centrale provenant de son site, au pied des hautes falaises de craie de la côte d'Albâtre, l'application de la loi Littoral doit être écartée pour ces travaux. Enfin, le texte supprime, à juste titre, la mise à l'arrêt définitif de plein droit d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner depuis plus de deux ans. L'actualité récente nous a montré que certaines centrales frappées par une longue mise à l'arrêt ont dû recourir à des dossiers de demande de dérogation chronophages et peu utiles. Ces mesures de simplification ont globalement été approuvées par la commission des affaires économiques, dont je salue l'esprit de responsabilité. Notre groupe proposera cependant quelques amendements de correction, visant à revenir sur des précisions qui ont été adoptées en commission et qui sont satisfaites par le code de l'environnement.

Hormis ces quelques points, nous nous félicitons qu'une grande partie des groupes politiques soutienne ce texte fondateur, première pierre d'un immense chantier pour la relance du nucléaire en France. Bien évidemment, notre groupe le votera. La parole est à M. Franck

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, parce que le Président de la République et les gouvernements qui se sont succédé depuis 2017 l'ont voulu ainsi, la question énergétique a été totalement absente du débat public pendant les cinq dernières années. Vous n'avez pas voulu aborder au fond cette question déterminante pour l'avenir de notre pays, madame la ministre. Et ce n'est pas faute de vous avoir souvent interpellée à ce sujet. Pourtant, les raisons ne manquaient pas : elles sont toutes liées à la question du changement climatique et à l'action immédiate qui en découle,

l'adaptation des modes de transport et de l'habitat, ou encore l'inflation, puisque l'énergie est au coeur de son mécanisme. Avant l'envolée des prix de l'énergie liée à la crise géopolitique en Europe, une crise de l'offre était déjà là.

Le quinquennat aurait dû être mis à profit pour engager la concertation avec les Français et le Parlement sur la stratégie sur l'énergie et le climat, préalable à la loi de programmation quinquennale et à la PPE qui en est la traduction opérationnelle.

La question n'est pas légère, et j'estime que le Parlement et les Français ont leur mot à dire. Aujourd'hui, en position de faiblesse et dans le cadre d'une logique qui défie le bon sens, vous nous demandez d'accélérer le développement des énergies renouvelables et vous nous proposez de simplifier, pour les quinze ans à venir, les procédures d'autorisation pour la construction de nouvelles installations nucléaires sur des sites existants ou à proximité immédiate. Ce que vous proposez permettra de gagner une année, voire deux, après en avoir perdu cinq, et ce pour des installations industrielles dont la durée de vie pourrait être de soixante ans ou plus. exprimé, on saisit mieux l'enjeu, qui, pour n'être pas du tout à la hauteur du sujet et de son urgence nationale, n'en est pas moins à considérer. Nous sommes globalement favorables à ces dispositions de simplification qui faciliteront le travail des opérateurs- EDF Production, RTE -et des filières industrielles concernées. Mais où le Président de la République et le Gouvernement veulent-ils amener le pays en matière de mix énergétique, Tous les réacteurs nucléaires anciens ne pourront être reconduits. Certains devront être mis à l'arrêt à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire- RTE l'a anticipé dans ses hypothèses d'études.

Nous proposerons des amendements de suppression de ces dispositions, car la PPE ne peut être traitée sur un coin de table, au détour d'un texte centré sur les procédures.

nous rappellerons que la loi doit garantir à EDF un caractère public d'entreprise intégrée, au coeur du futur énergétique de la Nation. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, août 2022 : par un projet de loi sur le pouvoir d'achat, le Gouvernement sécurise le relèvement du plafond de l'Arenh à 120

Texte après texte, la question de l'énergie est traitée segment par segment, petit morceau par petit morceau. Il est donc difficile d'entrevoir une cohérence ou une réflexion d'ensemble. Le sentiment qui prévaut est celui d'un traitement sur la forme, qui évite toujours les questions de fond. Qu'il s'agisse des énergies renouvelables ou du nucléaire, l'explication serait toujours la même : des procédures administratives trop longues, qu'il faudrait simplifier. La même recette se glisse dans tous les textes, saupoudrée d'un peu d'acceptabilité et de quelques mots magiques concertation, démocratie locale, discussion. Des points évidemment très importants, qui doivent être partie intégrante de la mise en pratique d'un texte. Mais pour qu'il y ait une mise en pratique,

Rien n'est dit sur le financement de ces nouveaux équipements. Votre texte n'en parle tout simplement pas. Qui va payer pour ces investissements ? EDF avec ses 60 milliards de dettes, dont une bonne partie vient de l'Arenh,

? Chaque fois que l'on pose la question, vous nous faites la même réponse, madame la ministre : « Les discussions sont en cours. » Cela veut bien dire que l'on réfléchit à créer des équipements, à investir, avant même de savoir comment on va exploiter la production. Rien ne justifie que l'État s'abstienne de mener une telle réflexion et, pourtant, silence radio dans votre texte- pas un mot. Autre point central : pourquoi la France construirait-elle de nouveaux réacteurs ? Pour sa souveraineté énergétique ? Pour son indépendance ? Pardonnez-moi, mais il n'y a aucune souveraineté possible avec le marché européen de l'énergie ! Vous payez pour la politique énergétique de vos voisins, que ces derniers cherchent ou non à sortir des énergies fossiles.

l'État veut détenir 100 % du capital. Très bien, mais pour quoi faire ? Pour bâtir un grand service public de l'énergie comme nous le souhaitons, ou pour scinder l'entreprise historique en plusieurs morceaux et l'ouvrir aux acteurs et aux capitaux privés ? Mystère ! On ne sait toujours pas, mais il faudrait voter un texte pour construire de nouveaux réacteurs, le tout alors que même le nouveau PDG d'EDF n'a pas encore défini sa feuille de route. En d'autres termes, nous n'avons même pas de visibilité sur l'existant, sur sa gestion, sur les ambitions, et même pas encore de PPE.

dont la durée de vie sera de soixante ans. L'urgence est donc non pas de réduire de quelques mois les procédures administratives sur des chantiers qui commenceront au mieux en 2027, mais bien d'avoir un débat politique et une vision de long terme. D'ailleurs- ce sera ma dernière question

c'est vous attaquer à toute la filière et lui faire perdre en attractivité. Comment allez-vous construire des réacteurs sans travailleurs et travailleuses qualifiés ? Si vous comptez sur de la sous-traitance en cascade, alors il faudra assumer que vous voulez du nucléaire et bas de gamme, avec des travailleurs précaires qui subiront votre réforme des retraites. C'est incompatible avec les enjeux de sûreté nucléaire. Votre texte vise à parler du nucléaire, mais sans parler du nucléaire.

L'atome doit être au coeur de notre politique énergétique. Plus qu'une conviction, c'est une certitude. Bienvenu et salutaire, ce projet de loi ne résout toutefois qu'une partie de l'équation posée par nos politiques énergétiques. Avec mes collègues du groupe Union Centriste, je regrette ainsi le désordre inhérent à l'examen parlementaire de notre politique énergétique. En décembre dernier, nous examinions le projet de loi d'accélération des EnR. Aujourd'hui, c'est le nucléaire. Et en juin prochain, dans le meilleur des cas, nous examinerons la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mes chers collègues, tout cela manque de lisibilité et de clarté. Nous devons pourtant poser les jalons d'une politique cohérente, afin de bâtir notre souveraineté énergétique à l'horizon 2050. Conçu comme un accélérateur, ce texte simplifie tant les procédures juridiques préalables à la construction des quatorze EPR, annoncée par le Président de la République lors de son discours de Belfort, que les contraintes pesant sur les sites existants. Il vise à réduire les freins, à lever les blocages et à contourner les obstacles qui condamnent aujourd'hui la construction des réacteurs et la modernisation des installations à une lenteur aussi désolante que problématique. Si le texte initial du Gouvernement allait dans le bon sens, je souhaite saluer le travail précieux des rapporteurs, Daniel Gremillet et Pascal Martin, ainsi que celui de la commission des affaires économiques et de la commission de l'aménagement du Ils rappellent tout l'intérêt de l'intervention parlementaire. Mes chers collègues, je souhaite que l'examen en séance publique nous permette de continuer d'enrichir le texte. À l'heure de la crise de l'énergie, il est de notre responsabilité de bâtir notre souveraineté en nous appuyant sur un mix énergétique décarboné,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, intervenant en treizième position dans cette discussion générale, après notamment les

Mes premiers mots seront pour le titre de ce projet de loi, censé traduire les intentions du Gouvernement. Permettez-moi, en tant que membre de la commission de la culture, d'en faire une présentation quelque peu iconoclaste, fondée sur plusieurs références culturelles bien connues du grand public, de manière à refléter le sentiment assez largement partagé. S'il fallait trouver un titre qui corresponde précisément aux objectifs affichés, j'opterais volontiers pour l'oeuvre de Marcel Proust,. C'est en effet parce que l'exécutif procrastine depuis dix ans sur la question du nucléaire que nous devons, en catastrophe, envisager les voies et moyens d'accélérer, afin de renouveler notre parc de réacteurs nucléaires. Dans cette assemblée, chacun sait que le temps perdu ne se rattrape pas. Je rappelle d'ailleurs que Proust a mis seize ans pour achever son oeuvre. Ma deuxième référence, empruntée cette fois au registre pictural, est, tant la gestion de la politique énergétique dans notre pays est un naufrage, dont les récentes tentatives de sauvetage relèvent davantage de la panique générale que d'un plan bien établi. troisième référence est la chanson de Dalida,, particulièrement appropriée pour décrire les déclarations successives du président Macron depuis deux ans, à grand renfort de communication, sans qu'aucune décision concrète soit venue les traduire de manière formelle à ce jour. Enfin, le populaire film synthétise bien les atermoiements que nous observons depuis 2017, notamment la valse des ministres qui se sont succédé à la transition écologique et énergétique, capables de dire tout et son contraire dans un laps de temps assez réduit. Le bilan du président Macron est lourd : deux pas en arrière avec la fermeture effective des deux réacteurs de Fessenheim, un bond dans le passé avec l'arrêt du programme de recherche Astrid sur les réacteurs de quatrième génération et, aujourd'hui, un tout petit pas en avant avec ce texte aux promesses bien ténues, portant essentiellement sur l'allègement des formalités administratives. Madame la ministre, le propos peut paraître quelque peu acide, mais il est temps de prendre des positions qui engagent de nouveau notre pays sur la voie d'une souveraineté que d'autres- le général de Gaulle et le président Pompidou en tête -ont su patiemment bâtir en assurant la construction de notre parc électronucléaire en moins de vingt ans. Une doxa idéologique s'est progressivement imposée dans le débat public national, appuyée par une communication- il faut le dire -assez efficace.

Il s'agit d'une légende urbaine couramment reprise jusqu'au plus haut niveau de l'État et dont le seul objectif est de discréditer la filière. filière. Pis, nous sommes aujourd'hui en infraction par rapport à notre propre législation, qui prévoit depuis 2006 la fermeture du cycle du combustible, que seuls les réacteurs à neutrons rapides permettent. Diviser par dix la quantité de déchets produits, limiter la prolifération de plutonium, pouvoir utiliser les 300 000 tonnes d'uranium appauvri disponibles sur notre sol, assurer la production d'électricité pour plus de 1 000 ans la promesse d'un nucléaire durable était trop belle et trop tangible pour que quelques idéologues ne nous empêchent pas habilement d'y accéder. On ne dira jamais assez à quel point l'arrêt du programme Astrid, en 2019,

Pour être encore plus clair, nous avons accepté quantité de mesures, louables au demeurant, visant à mettre fin au recours aux énergies fossiles, mais sans aucune mesure anticipant la tension que cela induirait sur la demande en électricité. Pis, les décisions visant depuis vingt-cinq ans à condamner la production d'origine nucléaire sur l'autel de petits arrangements politiciens nous ont conduits dans une impasse. Au bout de cette impasse,

Au pays des Lumières, notre destin énergétique est désormais entre les mains du gouvernement de l'ombre, qui tente de gérer la pénurie qu'il a lui-même organisée. Pour citer Bossuet, « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes Je salue pour terminer l'excellent travail, très approfondi, de nos rapporteurs pour pousser le curseur aussi loin que possible de manière à affirmer clairement de nouvelles ambitions pour notre pays. Madame la ministre, vos déclarations récentes laissent toutefois assez peu d'espoir quant à une position favorable du Gouvernement sur les grands principes plusieurs fois évoqués dans ce débat : revenir sur le plafond des 50 % de nucléaire dans notre mix électrique, prolonger, avec l'avis de l'ASN,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre vigilance est aujourd'hui appelée sur ce texte technique relatif à l'accélération du nucléaire français.

grande loi structurante de stratégie énergétique devrait être examinée par le Parlement au second semestre 2023, accélérer des

Du point de vue de l'aménagement du territoire, compléter des installations nucléaires ou créer de nouveaux EPR n'est pas neutre. Ces constructions peuvent-elles être pensées sans concertation dans un débat de techniciens, comme dans les années 1970 ?

L'acceptabilité sociétale du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle implique aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique, dans un contexte de transition et de décarbonation de notre économie. Ce texte qui vise à accélérer les procédures pour amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires ne devrait en aucun cas servir de support pour anticiper la future grande loi qui définira la stratégie française au long cours relative à l'énergie, au climat et à la composition de notre mix énergétique,

seront soumises ces nouvelles installations. La construction des six EPR qui seront encore en fonctions à l'horizon 2081-2090 effet l'évaluation des conditions climatiques locales dans lesquelles ces centrales vont fonctionner. Il s'agit notamment de mettre en oeuvre des études de descente d'échelle dynamique, absolument nécessaires en sus des éléments de projection globale issus Enfin, le nucléaire n'est pas seulement une question de normes. Il s'agit de donner du sens à ceux qui auront un réacteur près de chez eux, aux futurs personnels qui vont construire ces équipements, aux ingénieurs chargés de la sûreté de ces derniers, aux élus et à tous les acteurs, afin de mettre en évidence le sens profond des actions menées, qui manque aujourd'hui à beaucoup de citoyens.

le projet de loi que nous examinons aujourd'hui a pour objectif de faciliter le développement de l'énergie nucléaire au travers de la construction de nouvelles installations. La stratégie énergétique de la France n'a pas toujours été celle du nucléaire. En témoignent la fermeture de la centrale de Fessenheim en 2020 et celle, annoncée en 2018, de quatorze réacteurs d'ici à 2035. En témoignent également les propos d'une ancienne ministre de la transition écologique et numéro deux du Gouvernement qui jugeait en 2018 « absurde » la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et qui affirmait promptement « ne pas voir le nucléaire comme une énergie d'avenir ». Les temps ont donc changé, mais, comme le disait Edgar Faure, sans référence d'ailleurs à l'énergie éolienne : « Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent» De fait, la météo géopolitique, dorénavant plus imprévisible que la météo climatique, nous contraint à faire évoluer nos logiciels politiques. Nous avions un logiciel binaire, qui opposait, au fond, le nucléaire au renouvelable, considérant que l'un devait progresser au détriment de l'autre. Nécessité faisant loi, nous changeons de paradigme, forts de la conviction nouvelle que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais bel et bien l'un et l'autre- Sophie Primas l'a fort bien indiqué dans son intervention. Piégés par ce pseudo-dogme qui s'est traduit par des volte-face, nous avons perdu beaucoup de temps, car, après avoir facilité la destruction, nous facilitons dorénavant la construction. Le nucléaire, qui n'est pas exempt de défauts, fournit d'indéniables réponses aux problèmes climato-géopolitiques du moment : il est décarboné, sa capacité de production est modulable et adaptable aux besoins de la population et, surtout, il est synonyme d'indépendance énergétique et, partant, diplomatique et politique. La recherche gomme d'ailleurs au fur et à mesure les défauts de cette technologie. Les récentes découvertes scientifiques californiennes dans le domaine de la fusion nucléaire, singulièrement la capacité à franchir le seuil d'ignition, c'est-à-dire le stade où les réacteurs produisent davantage d'énergie qu'ils n'en consomment, sont particulièrement prometteuses. certes beaucoup de temps, mais à l'évidence, les innovations attendues nous amèneront probablement à porter un autre regard sur ce mode de Ce projet de loi permet donc d'accélérer la construction de nouveaux réacteurs en France, d'une part, en simplifiant les différentes procédures urbanistiques ou environnementales, et, d'autre part, en clarifiant les modalités de réexamen périodique des réacteurs de plus de C'est un premier pas. L'article 1 délimite le champ d'application de ce texte aux constructions jouxtant les parcs nucléaires existants, comme celui de Penly, près de Dieppe, que j'ai d'ailleurs visité avec notre collègue et rapporteur pour avis Pascal Martin. L'avenir, « plus difficile à prévoir que le passé », comme dirait Woody Allen, nous imposera probablement d'élargir le champ des possibles par la construction de petits réacteurs- les fameux SMR -capables de fournir des solutions dans les sites isolés. les sites isolés. Cette stratégie d'ensemble doit être pensée sur le temps long, comme cela a d'ailleurs été rappelé en commission, et elle devra englober à la fois l'amont, avec l'approvisionnement en combustible et les ressources en uranium, et l'aval, au travers de la nécessaire question de la gestion des déchets. Nous devons également soutenir la formation, le recrutement et la recherche dans le domaine du nucléaire. Autrefois perçu comme une filière d'excellence, le nucléaire est aujourd'hui confronté à une réelle pénurie de talents. Face aux tergiversations politiques, nos jeunes ingénieurs et techniciens se sont détournés depuis longtemps du nucléaire, lui préférant d'autres industries plus pérennes, quand ce ne sont pas les cabinets de conseil. Il est crucial de renforcer l'attractivité de la filière, la formation de personnels qualifiés étant la clé d'une filière industrielle solide. C'est donc un grand chantier national, ... Veuillez

des décisions qui pourraient être prises sur la production nucléaire, et pour accélérer la production d'énergies renouvelables- vous le savez comme moi, nous sommes déjà en retard sur les objectifs de production renouvelable pour les années 2018-2023.

En 2019, nous signions un contrat stratégique de filière nucléaire, qui programmait notamment le renforcement des compétences et le renforcement de la sous-traitance. En 2020, c'était l'un des six secteurs prioritaires mis en avant dans le cadre du plan de relance, avec un plan de montée en en investissement de 472 millions d'euros pour les sous-traitants de la filière nucléaire. En 2021, nous lancions France 2030, avec 1,2 milliard d'euros pour la recherche et développement, ainsi que l'innovation, qui s'ajoutent aux montants déjà existants.

au renforcement des compétences, ce qui conduit à prendre des décisions sur le territoire- je pense notamment à la région Normandie. En 2022, nous avons engagé les débats sur le mix énergétique

de façon à mettre en accord nos paroles et nos actes, nous ne reviendrons pas sur la modification apportée en commission au plafond

l'exposé des motifs du projet de loi que nous examinons insiste sur « notre besoin impératif et souverain d'indépendance énergétique ». Cette ambition de l'indépendance énergétique de la France affichée par le Gouvernement justifie une mise en cohérence avec l'arrêt des exportations d'uranium de retraitement à l'étranger. Les conditions environnementales et de stockage en Sibérie, à Tomsk, n'ont jamais été rendues publiques, et les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'en assurer. Le Gouvernement a par ailleurs demandé aux industriels du secteur nucléaire de mettre un terme à leurs exportations d'uranium de retraitement vers la Russie. Cela a notamment été confirmé par l'Association nationale des comités et commissions locales d'information, lors d'une réunion du 18 novembre 2022 au cours de laquelle la société EDF a fait état de cette demande.

la France est tributaire de nombreux pays, dans l'ordre le Kazakhstan, l'Australie, le Niger et l'Ouzbékistan, ainsi que la Russie, pour enrichir l'uranium naturel. Entre 2000 et 2012, elle a importé de Russie près de 1 000 tonnes d'uranium enrichi par an, soit presque la totalité de sa consommation. On n'en parle pas beaucoup ... Sur les neuf premiers mois de 2022, malgré la guerre en Ukraine, la France a importé 290 tonnes d'uranium enrichi de Russie, près du tiers de sa consommation Orano précise que près de 44 % des ressources en uranium se situent dans les pays de l'OCDE, ce qui mettrait les importations à l'abri de chantages géopolitiques. C'est moins évident pour les filières d'enrichissement. Les importations se font au prix de compromissions avec certains régimes autoritaires, et au mépris de la santé des populations locales. L'ambition de sécurité de l'approvisionnement et la question de la fiabilité des partenaires commerciaux- un risque géopolitique élevé dans le secteur du nucléaire -commandent une nécessaire transparence de l'État et des acteurs industriels français. C'est pourquoi nous proposons la publication, par les exploitants publics et privés, d'un rapport annuel sur les importations et les exportations d'uranium. Un peu de transparence ne nuit pas ...

dans le cadre des procédures de participation du public, le code de l'environnement exclut la divulgation d'éléments de nature à porter atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique et des personnes et à la conduite de la politique extérieure de la France, ainsi qu'au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pénales et aux droits de propriété intellectuelle. Demande de retrait

Non, je ne confonds pas souveraineté, indépendance et sécurité. Il est faux de dire que, sur le nucléaire, nous sommes souverains, parce que nous dépendons de l'uranium kazakh, russe ou nigérien, extrait dans de mauvaises conditions sociales et environnementales. Oui, il faut le dire.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en tant que sénatrice alsacienne, je ne peux que regretter les décisions prises depuis une dizaine d'années sur les centrales nucléaires, et particulièrement celle de Fessenheim, qui aurait pu être maintenue en activité si nous n'avions pas fait le choix de sacrifier la souveraineté énergétique française aux intérêts économiques et politiques de nos voisins allemands.

peu de temps avant sa fermeture, pour la maintenir au plus haut niveau, et qu'en dépendaient 3 000 emplois directs et indirects. Pour compenser les pertes d'activité et d'emplois, et pour rendre cette décision acceptable auprès des habitants et des élus locaux, un projet franco-allemand a été sorti du chapeau, dans l'urgence. Une société d'économie mixte a été créée, sans anticipation ni réflexion, ce qui s'est soldé par un échec : elle a été dissoute sans avoir mené un seul projet et après avoir coûté 1 million d'euros. Enfin, les projets annoncés de reconversion du site, dont le fameux technocentre d'EDF, et pour lesquels le Président de la République a promis 20 millions d'euros dans son discours de Belfort du 10 février 2022, sont restés bloqués au stade de l'affichage. Qu'en est-il, madame la ministre ? Au moment où vous envisagez la fermeture d'autres sites nucléaires, le cas de Fessenheim a de quoi nous inquiéter. Des élus locaux n'ont pas été écoutés, les habitants ont été méprisés et les promesses n'ont pas été honorées. Je me félicite que le texte du Sénat s'inscrive enfin dans une stratégie globale, avec des perspectives de planification, afin de ne pas reproduire de telles décisions brutales, incohérentes et contraires aux intérêts des territoires. La parole est à M. François Bonhomme, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, on peut toujours dire qu'il ne s'agit, avec ce texte, que de débroussailler le terrain administratif et juridique en attendant une feuille de route et la relance formelle du nucléaire, avec des centrales de nouvelle génération et la reconstitution d'un parc performant. Toutefois, madame la ministre, à ce

quand on se laisse intoxiquer, dans tous les sens du terme, par une Allemagne qui nous fait la leçon tout en laissant tourner à plein ses centrales à charbon. Ce texte est la première étape d'un revirement que vous vous obstinez encore à qualifier d'anticipation et d'accélération, comme si ce n'était qu'un changement de rythme, alors que nous devons prendre une nouvelle orientation. Vous faites mine de découvrir que la production d'électricité nucléaire doit être la colonne vertébrale de notre modèle énergétique. Pourtant, les conséquences d'aujourd'hui découlent en grande partie de vos choix passés de notre capacité de production énergétique, faisant de notre pays, pour la première fois, un importateur net d'électricité de nos voisins européens, produite avec du gaz et du charbon ; vulnérabilité structurelle de notre approvisionnement ; explosion des coûts subis par les collectivités, les ménages et les entreprises dépenses budgétaires considérables et, malgré tout, insuffisantes pour amortir le choc inflationniste ; enfin, dégradation de notre solde commercial. Et vous avez l'impudence, madame la ministre, de vous féliciter du succès de votre plan de sobriété ... Il faut beaucoup d'estomac pour l'affirmer.

même au nucléaire, et pas seulement de futures installations sur certains sites prédéfinis. Ce grand débat, à la mesure de ce que représente ce choix, stratégique et politique, reste selon moi le premier impératif.

terrible erreur attentant gravement à notre souveraineté énergétique, je voudrais juste rappeler quelques éléments. Ses deux réacteurs n'étaient manifestement pas en mesure de passer leur quatrième visite décennale (VD4), qui aurait dû intervenir en 2020 pour l'un et en 2022 pour l'autre.

L'ASN a donc accordé un délai supplémentaire, mais, sous prétexte de fermeture de la centrale, EDF a refusé cette prescription. Le renforcement du radier séparant les réacteurs de la nappe phréatique avait été très insuffisant

la falsification commise aux ateliers du Creusot pour faire passer des aciers non conformes- on se souvient des fameux dossiers barrés -a touché de nombreuses centrales : à Fessenheim, la virole, qu'il avait fallu remplacer sur le générateur de vapeur n° 335,

réacteurs étaient en fin de vie et, par pragmatisme, les investissements pour se hisser au niveau requis pour la VD4 n'avaient pas été jugés possibles. La

avec les ingénieurs, les syndicats, mais également les responsables d'EDF, tous nous disent que la question de la sous-traitance est posée en grand.

la relance du programme nucléaire national. Je ne vous apprends normalement rien en le disant. Décider de manière cavalière, unilatérale et antidémocratique le remplacement de l'objectif de réduction de 50 % de l'énergie nucléaire d'ici à 2035 par un objectif de maintien à 50 % au moins de cette énergie à l'horizon 2050, pour relancer la filière nucléaire, ou encore l'introduction d'un objectif de production d'énergie nucléaire à partir de matières recyclées- de 20 % d'ici à 2030 -pour valoriser le cycle du combustible n'est pas opportun, alors que le débat public sur les EPR 2 est en cours, et ce jusqu'à fin février, et que la concertation publique sur le mix énergétique n'a pas encore eu lieu. Ces nouveaux objectifs sont définis de manière prématurée. Toutes les garanties doivent être apportées pour que les décisions politiques soient prises dans le respect du Parlement et de nos concitoyens, ce qui n'a pas l'air d'être facile quand il s'agit du nucléaire ... Tout cela ne doit pas être décidé unilatéralement et en catimini. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. La

Je veux simplement rappeler l'enjeu démocratique que représente la possibilité pour les Français de s'exprimer sur la question de la politique énergétique de leur pays. Il s'agit d'une exigence constitutionnelle,

qu'il fallait marcher sur nos deux jambes, le nucléaire et les énergies renouvelables. Cela nous renforce dans notre conviction

parfois même à leur corps défendant, à aborder les débats sous un angle idéologique. Or, si nous avons besoin d'un mix énergétique, cela n'est pas d'abord pour des raisons idéologiques,

Merci

ouvrons aujourd'hui et publiquement, avec le soutien de ceux qui proposent un texte- la commission -et avec l'apport utile de ceux qui le combattent, un débat qui obligera

Merci

existant. Il nous faudra plusieurs décennies pour nous en affranchir, mais il est primordial de ne pas relancer du « nouveau » nucléaire. Nous souhaitons donc sécuriser le cadre juridique en vigueur, en rappelant que tout projet de réacteur nucléaire supplémentaire doit demeurer cohérent avec le mix énergétique et avec l'obligation de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. C'est tout le débat que nous avons en ce moment. Nous ne partageons pas votre vision, encore l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Aujourd'hui, seul l'exploitant a la possibilité de demander l'abrogation des autorisations d'exploiter lorsque le plafond de 63,2 gigawatts est susceptible d'être dépassé. ce plafond a pour seul objectif d'éviter l'extension du parc nucléaire et ne permet pas de remplir les objectifs de réduction de la part du nucléaire fixé par la loi. Ainsi, en donnant au ministre chargé de l'énergie le pouvoir de fermer les centrales nucléaires, nous souhaitons éviter de faire reposer entre les mains exclusives de l'exploitant la possibilité d'abroger des autorisations d'exploiter et garantir le respect des objectifs de décarbonation du mix et de réduction de la part du nucléaire. Ce n'est pas à l'exploitant de piloter la politique énergétique française ... Quel est l'avis de la commission ? Madame la ministre,

la politique énergétique en matière de production d'électricité d'origine nucléaire ont été complétés pour tenir compte de la construction de six, voire de quatorze EPR supplémentaires annoncée par le Gouvernement. B nouveau prévoit en particulier de recourir à une part de 20 % de matières recyclées dans la production d'électricité nucléaire à l'horizon 2030, à des fins de valorisation du cycle du combustible. Une telle voie est souhaitable, car elle peut

-seront précisées dans la future loi quinquennale sur l'énergie. Encore une fois, ce maximalisme en matière de relance du nucléaire, très engageant pour nos choix énergétiques stratégiques, met les parties prenantes et l'ensemble de nos concitoyens devant le fait accompli.

portant sur l'effort budgétaire afférent à la sûreté, à la sécurité, à la recherche, à l'innovation ou encore au recyclage et au stockage des déchets. En outre,

EDF envisage actuellement de construire une première paire de nouveaux réacteurs sur le site de Penly, en Normandie, une deuxième paire sur le site de Gravelines, dans les Hauts-de-France, puis une troisième paire sur un site nucléaire existant dans la vallée du Rhône- Bugey ou Tricastin. Dans le cadre du débat public en cours, EDF a préparé un dossier complet sur les enjeux du programme, qui est disponible sur le site de la Commission nationale du débat public. Comme l'a demandé le EDF a engagé, depuis février 2022, des études pour huit réacteurs EPR 2 supplémentaires, sans conclusion à ce stade en matière de calendrier ou de localisation, et ce travail doit se poursuivre dans les meilleures conditions, afin qu'une proposition industrielle puisse émerger. En réponse aux attentes exprimées par les parlementaires, le Gouvernement propose de transmettre au Parlement, avant la discussion de la loi de programmation relative à l'énergie et au climat prévue en 2023,

D'autre part, point également très important, les éléments évalués seraient moins nombreux, puisqu'ils ne viseraient plus la situation du groupe EDF, du marché de l'électricité et des finances publiques.

mais qui sont de nature à répondre aux questions émergeant dans le débat public sur le nouveau programme nucléaire et qui éclaireront le débat parlementaire. Par cet amendement, il s'agit d'évaluer également l'impact sur l'ensemble du cycle du combustible de l'amont à l'aval, notamment sur l'approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, ainsi que sur la revalorisation du combustible usé. les réserves mondiales d'uranium exploitable représenteraient plus d'un siècle d'exploitation au rythme actuel, mais on ne peut présager des difficultés d'approvisionnement en cas de relance ambitieuse du nucléaire au niveau mondial et de conflits géopolitiques. Le rapport de RTE, publié avant le conflit en Ukraine, l'a souligné : « La disponibilité des réserves d'uranium naturel à long terme fait aujourd'hui l'objet de moins d'inquiétude, dans un contexte où de nombreux pays prévoient de fermer leur parc de réacteurs nucléaires et où le nombre de réacteurs en construction reste limité. » Depuis lors, les cartes ont été rebattues et le regain d'intérêt pour le nucléaire en France et à l'international risque de rendre obsolètes les hypothèses des différentes projections. D'où la nécessité de compléter l'article 1D par le présent amendement. Quel

Assemblée, dans la mesure où la notion de cycle de combustible englobe déjà les enjeux de l'approvisionnement en uranium et la revalorisation du combustible usé. Ainsi, cet amendement est déjà satisfait sur le fond par la rédaction actuelle.

du marché de l'électricité et des finances publiques devienne peu à peu une préoccupation. De notre côté, nous devinons déjà la conclusion de ce rapport : la situation d'EDF est catastrophique et il est urgent d'intervenir. Comme nous l'avons déjà dit, nous regrettons que rien ne soit prévu dans ce texte pour corriger le tir contre la mise en concurrence et contre l'Arenh, qui sont responsables de la situation d'EDF et des prix exorbitants de l'énergie. Par cet amendement, nous souhaitons alimenter la réflexion sur le nucléaire. Nous partageons en effet certaines préoccupations portant notamment sur le traitement des déchets. Si la plupart des modes de production d'énergie engendrent des déchets, ceux du nucléaire ont la particularité d'être radioactifs et de mettre, pour certains, des dizaines de milliers d'années à disparaître. S'il y a eu d'importants progrès concernant le recyclage, mais aussi la capacité à réduire la production des déchets, notamment avec les EPR de dernière génération, nous proposons de poursuivre ce travail de recherche sur les déchets, à la fois pour pérenniser l'énergie nucléaire et pour la rendre plus sûre au regard de notre environnement et de notre santé.

qui, ne l'oublions pas, fonctionneront encore à l'horizon 2080, doit prendre en compte les conditions climatiques locales dans lesquelles ils fonctionneront. Il s'agit notamment de mettre en oeuvre des études de descente d'échelle dynamique, absolument nécessaires, outre les éléments de projection globale du Giec. En termes de sûreté nucléaire, la connaissance exacte des événements environnementaux locaux est indispensable. Il s'agit par exemple, pour les installations sur le Rhône, de mieux anticiper l'hydrométrie du fleuve, ses évolutions de température, les phénomènes climatiques qui se développeraient notamment autour des sites nucléaires. D'après les données du Giec,

À l'horizon 2080, les débits du Rhône pourraient être profondément modifiés. Les études de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la Compagnie nationale du Rhône vont dans le même sens. Certains projets de recherches ont abouti à la création de scénarios climatiques régionalisés sur un ou plusieurs bassins versants incluant le territoire Rhône-Méditerranée. Ces données sont

doivent demeurer exceptionnelles et limitées dans le temps, nous souhaitons restreindre le champ d'application du titre I aux seuls six EPR 2 dont la construction a été annoncée par le Président de la République dans son discours de Belfort. Nous plaidons pour une accélération des procédures afin de consolider rapidement notre mix énergétique et d'éviter tout risque de rupture de notre système électrique, par exemple face à une situation de froid extrême. Si ce projet de loi est un texte d'anticipation destiné à amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, les mesures d'anticipation ne doivent toutefois pas devenir la règle.

de la loi, de tout un arsenal de mesures de simplification et d'accélération permettant d'amorcer la relance du nucléaire. En parallèle

disposerons donc d'une feuille de route qui devrait permettre de basculer de nouveau dans les procédures normales de droit commun. Tel est l'objet de cet amendement, qu'il faut voir comme un amendement de compromis, madame la ministre.